monsieur le ministre,

d'actes de terrorisme et au renseignement, et au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et du projet de loi de finances rectificative pour 2021 ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour l'examen du projet de loi de finances rectificative

a été largement mobilisé. Cela nous a amenés à utiliser la trésorerie disponible sur l'activité partielle de longue durée, comme c'était prévu dans le cadre du plan de relance. Le crédit de 6,4 milliards d'euros que nous vous proposons d'ouvrir permet donc à la fois de financer

Nous souhaitons aussi inscrire 150 millions d'euros de mesures spécifiques et sectorielles pour la culture, afin d'accompagner la sortie de crise du secteur, qui a connu, vous le savez, des difficultés. Et nous vous proposons- j'y reviendrai dans un instant -d'inscrire 200 millions d'euros de soutien aux collectivités locales, en particulier à celles qui gèrent un certain nombre de services publics en régie et qui ont vu leurs recettes très largement détériorées par la crise économique. Ces 15,5 milliards d'euros de mesures d'urgence représentent un engagement massif de l'État et expliquent la dégradation du déficit, sur laquelle je reviendrai à la fin de mon propos.

voulons aussi permettre des redéploiements pour assurer le financement des dispositifs relatifs à l'industrie du futur, mais aussi à la numérisation de l'économie et à l'agriculture. Autant de dispositifs qui ont connu un succès plus important que nous ne l'avions prévu et qui nécessitent de voir les crédits qui leur sont affectés rehaussés.

autres, par des annulations de crédits placés en réserve de précaution. Nous avons fait en sorte de ne jamais annuler plus de 30 % à 40 % d'une même réserve de précaution.

sera moins importante que prévu. D'autre part, nous avons permis aux entreprises de reporter la date de première échéance de remboursement, ce qui éloigne mécaniquement le risque de sinistralité. Si les mesures que nous vous proposons d'inscrire ne dégradent pas le déficit public, elles permettent de consacrer 700 millions d'euros à l'hébergement d'urgence : nous avons pris la décision de maintenir le nombre de places pendant tout l'été au même niveau que pendant la période hivernale. hivernale. En outre, 350 millions d'euros sont inscrits au bénéfice de l'agriculture pour financer les premières mesures d'indemnisation des agriculteurs touchés par le gel au cours du printemps dernier, mais aussi pour assurer le financement de dispositifs spécifiques, notamment en matière de grippe aviaire ou de jaunisse de la betterave. Il s'agit aussi de financer le Pass'Sport, annoncé par le Président de la République, à hauteur de 100 millions d'euros ; de mettre en place des mesures spécifiques aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour 57 millions d'euros d'assurer le financement de l'augmentation des bourses versées aux étudiants du fait de la dégradation de la situation économique l'année dernière, à hauteur de 150 millions d'euros ; et, enfin, de prévoir une aide spécifique à la Nouvelle-Calédonie, pour 82 millions d'euros.

de lettres », tendant notamment à reconduire pour la troisième année consécutive la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, exonérée de fiscalité et de cotisations. Cette prime exceptionnelle, que les entreprises peuvent verser si elles le veulent, a bénéficié à 3,1 millions de personnes l'année dernière au sein de 560 000 établissements. Nous avons jugé utile de la reconduire pour permettre aux entreprises le souhaitant et le pouvant d'accompagner et de reconnaître l'investissement de leurs salariés.

Il s'agit d'indemniser les régies, qui, confrontées à des situations souvent très particulières, ont connu une année 2020 extrêmement difficile. Il s'agit en général de régies présentant une forme d'asymétrie dans leur organisation, avec des services publics administratifs assurés par des agents recrutés avec des contrats de droit privé ou, au contraire, des services publics industriels et commerciaux assurés par des agents recrutés avec des contrats de droit public ou dans le cadre du statut de la fonction publique. ces raisons, ces régies ont pu perdre beaucoup de recettes tarifaires sans pouvoir bénéficier des dispositifs d'accompagnement propres au secteur concurrentiel comme le prêt garanti par l'État, la mise en place de l'activité partielle ou encore le fonds de solidarité. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un dispositif qui autorisera la compensation de la perte d'épargne brute de ces régies à hauteur de 120 millions d'euros. Nous avons veillé à faire en sorte qu'il concerne à la fois les communes, les intercommunalités, mais aussi leurs établissements publics. publics. Un certain nombre de délégations de service public pourront être intégrées, dans des cas très particuliers, à ce dispositif de soutien. J'aurai l'occasion de vous présenter un amendement

Il y a dans le dispositif propre aux collectivités locales une deuxième enveloppe de 80 millions d'euros. Elle a pour objet d'accompagner les collectivités, communes et intercommunalités, qui, du fait d'une perte de recettes tarifaires plus importante que la moyenne, auraient vu leur épargne brute chuter de manière extrêmement importante, en tout cas beaucoup plus fortement que la baisse d'épargne brute des communes et des intercommunalités, une baisse que nous estimons à 7,5 % pour l'année 2020. Ces mêmes dispositions « de lettres » permettront un certain nombre d'avancées. Elles sont le fruit d'amendements déposés par les députés et adoptés par l'Assemblée nationale.

qui le porte à 3 milliards d'euros. Ainsi, les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie, des difficultés de liquidité ou de fonds propres, confrontées au refus ou à une impossibilité d'accompagnement du secteur bancaire, alors même qu'elles interviennent dans un secteur viable ou connaissent des difficultés conjoncturelles, pourront être accompagnées par l'État dans le cadre de prêts de longue durée leur permettant de traverser la reprise d'activité, donc de faire face à la crise. De telles dispositions ont évidemment des conséquences.

a considéré que la récession connue en 2020 n'était pas de 8,2 %, mais de 7,9 %- je rappelle que nous avions travaillé aussi sur des hypothèses à 11 %.

Nous aurons, dans les temps à venir, et notamment lors de l'examen du projet de loi de finances, à souligner un certain nombre de nécessités : revenir à un niveau plus soutenable de dépenses publiques publiques ; veiller à ce que les mesures d'urgence et de relance que nous avons mises en place gardent un caractère ponctuel, circonscrit dans le temps et dans l'espace pour ne pas entraîner une augmentation trop importante du poids de la dépense publique et obérer ainsi nos capacités de rebond

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'encre du décret d'avance par lequel le Gouvernement prévoyait l'ouverture et l'annulation de crédits à hauteur de 7,2 milliards d'euros n'était pas encore sèche que l'on nous annonçait le dépôt, quelques jours plus tard seulement, d'un projet de loi de finances rectificative ! Nous voilà réunis pour l'examiner. Sur la forme, comme vous le savez, monsieur le ministre, j'étais partisan du dépôt plus précoce d'un texte devant le Parlement, dès le mois de mai, permettant tout de suite un examen par les deux assemblées et une discussion sur les mesures proposées par le Gouvernement. Tous, nous espérons que ce texte sera bien celui de la sortie de crise avec un soutien en faveur des entreprises encore touchées par les dernières contraintes et une pleine mise en oeuvre du plan de relance. Malheureusement, les nouvelles du front sanitaire entament un peu notre optimisme des dernières semaines. Du point de vue macroéconomique, avec un taux de 5 %, l'hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement apparaît- il faut le dire -raisonnable. Mais ne nous réjouissons pas trop tôt : le rebond d'activité demeure fragile et devrait être moins important que celui de nos principaux partenaires européens.

Ce qui mérite également de nous alerter et nous engage collectivement pour l'avenir est la très forte dégradation de nos finances publiques, avec un déficit de 9,4 % du PIB. Cette dégradation par rapport à la loi de finances initiale s'élève en valeur à près de 34 milliards d'euros. Ce sont principalement les hausses de dépenses liées à la crise qui l'expliquent. Sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », les ouvertures de crédit du PLFR sont de 9,8 milliards On nous demande d'ailleurs des rallonges budgétaires, notamment sur le fonds de solidarité, alors que le Gouvernement n'a pas encore clairement indiqué quelles seraient les modalités retenues pour les prochains mois. Je compte sur vous pour nous en dire plus, 2 milliards d'euros sont ouverts au titre des participations financières de l'État alors que des crédits avaient été annulés dans le décret d'avance quelques jours auparavant. Le déficit budgétaire de l'État s'élève à lui seul à 220 milliards d'euros. Ce montant, s'il est effectif, constituera de loin le déficit budgétaire le plus important jamais connu, y compris en incluant 2020. Pour autant, la dégradation du solde public apparaît presque sans effet sur le montant de la dette, dont le volume diminuerait par ailleurs, pour s'établir à 117,2 % du PIB. À court terme, et en sortie de crise, une telle situation se comprend. En revanche, il est indispensable que la France s'inscrive à compter de 2023 dans une trajectoire de réduction des déficits, comme le prévoit d'ailleurs le programme de stabilité.

Au demeurant, nos partenaires européens devraient, eux, retrouver une maîtrise de leurs comptes publics bien plus rapidement que la France. Il y va donc aussi de la crédibilité de notre pays sur les marchés financiers ; ne l'oublions pas. Les efforts devront être réalisés en intervenant sur les dépenses publiques.

À ce titre, monsieur le ministre, je réitère mon scepticisme face à l'inventivité de votre ministère concernant ces reports, qui atteignent un niveau exceptionnel cette année et vont, à mon sens, bien au-delà de l'autorisation parlementaire. Par ailleurs, l'augmentation des dépenses répond à un motif de précaution et d'extrême prudence qui va au-delà du nécessaire soutien à l'économie en période de crise. En effet, les montants inscrits au titre des différentes mesures de soutien restant actives se révèlent particulièrement élevés. C'est pourquoi il nous semble exagéré que le Gouvernement demande parallèlement l'alimentation à hauteur de 1,5 milliard d'euros de l'enveloppe des « dépenses accidentelles et imprévisibles ». Nous proposerons de la réduire à 500 millions d'euros. De surcroît, le Parlement ne saura qu'comment ces crédits seront utilisés. Cela donne l'impression de « chèques en blanc » faits au Gouvernement alors que de nombreux reports et mouvements budgétaires ont déjà été opérés.

Dans le même ordre d'idées, nous vous proposons de prolonger sur 2021 l'obligation pour le ministre de l'économie de nous informer avant toute opération réalisée sur des crédits ouverts sur le budget général au titre des participations financières de l'État. En principe, ce PLFR doit aussi s'inscrire dans la concrétisation de l'accélération de la mise en oeuvre du plan de relance. Or la consommation des crédits alloués reste encore très limitée avec, pour la mission « Plan de relance », 3,8 milliards d'euros de crédits de paiement décaissés, si l'on exclut les dépenses liées à l'activité partielle d'urgence, soit un taux d'exécution de seulement 18,1 % au bout d'un semestre. Plusieurs autres postes de dépenses publiques doivent également être surveillés de près. Sur l'hébergement d'urgence, l'abondement prévu de 700 millions d'euros est très important, mais peut-être insuffisant au regard des besoins que le rapporteur spécial Philippe Dallier a précisément décrits dans un récent rapport de contrôle sur le sujet. De même, le monde agricole a subi plusieurs crises cette année, notamment un épisode de gel tardif et une nouvelle épidémie de grippe aviaire. Le projet de loi de finances rectificative ouvre 350 millions d'euros, quand le Gouvernement a annoncé 1 milliard d'euros destinés aux seuls agriculteurs victimes du gel tardif. Même si certains crédits n'auront à être ouverts qu'en fin d'année, nous proposons un amendement de crédit pour rehausser ce montant dès la présente

De même, la commission des finances soutient la prolongation de l'octroi de garantie de l'État au titre des PGE, ainsi que la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Nous pensons toutefois nécessaire de permettre plus facilement aux entreprises de moins de cinquante salariés de verser une prime exonérée d'impôt et de prélèvements sociaux et allant jusqu'à 2 000 euros.

les députés sont revenus sur cette date, pourtant annoncée par le Gouvernement, en ne retenant en définitive que le 1 juillet 2022. Or il nous apparaît qu'il faut revenir avec pragmatisme sur une telle niche fiscale. Les secteurs concernés ont été durement touchés par la crise et les solutions de substitution à l'utilisation du gazole restent balbutiantes. Dans un souci de respect des engagements et d'équité entre les Français ayant permis à notre pays de tenir le choc au plus fort de la crise, la commission des finances vous propose également d'exonérer d'impôt sur le revenu la majoration exceptionnelle de l'indemnisation des internes. Si les praticiens hospitaliers ont pu en bénéficier pour la majoration de leur indemnisation, tel n'a pas été le cas des internes. monsieur le ministre, ces personnels ont été en première ligne pendant la crise sanitaire. Nous demandons au Gouvernement de tenir sa promesse. Plusieurs amendements s'inscrivent aussi dans la démarche de soutien à la reprise économique en complétant utilement les mesures déjà en vigueur ou dans le texte. Ainsi en est-il de la traduction dans notre législation d'un mécanisme fiscal de déduction pour le capital à risques, qui porte ses fruits chez certains de nos voisins européens qui est préconisé par le FMI et la Commission européenne. Il s'agit ainsi d'inciter à la levée de fonds propres, en neutralisant le biais fiscal en faveur de la dette. Un dispositif permet également d'encourager les entreprises à investir dans la transition écologique, même en temps de crise. Plusieurs mesures d'un coût modeste permettent aussi d'apporter un dernier soutien à certaines entreprises qui ont pu rencontrer des difficultés pour obtenir de l'aide ou qui sont particulièrement touchées par des crises sanitaires. Nous souhaitons également proroger jusqu'à la fin de l'année 2022 le relèvement à 1 000 euros du plafond des dons éligibles à la réduction d'impôt du dispositif dit Coluche pour soutenir le tissu associatif directement en contact avec les personnes défavorisées. Enfin, à propos des collectivités territoriales, il est proposé de reconduire en 2021 les « filets de sécurité » qui étaient prévus en 2020 pour certaines ressources spécifiques des collectivités d'outre-mer et de la collectivité de Corse, comme c'est le cas pour les autres dispositifs de droit commun. Mes chers collègues, avec ce texte, nous traitons aujourd'hui la sortie de crise avec un soutien à la reprise et à la relance. La majorité des amendements déposés ou soutenus par la commission iront dans ce sens. Une suppression « en sifflet » des mesures d'urgence adoptées pendant la crise, proportionnée en fonction des secteurs et de l'évolution de la reprise de leur activité, est nécessaire. Il faut sortir de l'économie « sous perfusion » des aides de l'État. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission des finances vous propose d'adopter ce projet de loi de finances rectificative

le 12 mai dernier, le Gouvernement soumettait aux commissions des finances un décret d'avance portant ouverture de 7,2 milliards d'euros afin d'abonder le fonds de solidarité pour les entreprises et de financer l'activité partielle, mais, dès le 2 juin, il est apparu que cette somme n'était pas suffisante au regard des besoins et que la présentation rapide d'un collectif budgétaire s'imposait. de finances rectificative, qui ouvre des crédits supplémentaires pour les dispositifs déjà cités, mais également pour quelques autres, comme l'hébergement d'urgence, le transport aérien ou le monde agricole. Les recettes sont par ailleurs très légèrement revues à la hausse. La principale information délivrée par ce texte réside moins dans ces mesures complémentaires que dans la réévaluation drastique du déficit attendu en fin d'année, puisqu'il bondirait de 178,1 milliards à 220 milliards d'euros, soit 9,4 % du PIB. Cette situation inédite n'est pas liée aux mesures nouvelles, mais principalement au volume de crédits reportés de 2020 sur 2021, presque 30 milliards d'euros. On peut tout aussi bien s'effrayer de ce nouveau déficit attendu que s'interroger sur la sincérité des prévisions d'exécution des crédits budgétaires, lorsque l'on remarque que seulement un cinquième des crédits du plan de relance a été consommé à la mi-juin, hors chômage partiel. Par ailleurs, le Gouvernement ne peut plus recourir à un décret d'avance, puisque les montants maximaux ont été utilisés par celui du 19 mai. Il propose donc de provisionner une dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles pour pouvoir ouvrir des crédits sans nouvel examen parlementaire. Certes, la crise conduit à devoir réagir rapidement, mais il importe que l'on ne demande pas au Parlement de signer des chèques en blanc pour couvrir toutes les hypothèses L'an passé, tous les crédits pour faire face à la crise ont été examinés par le Parlement, sous des contraintes finalement bien plus fortes. Au-delà de l'abondement du fonds de solidarité, le texte présente d'autres points positifs comme le soutien à certaines régies publiques locales ayant subi des pertes tarifaires- nous demandons cette mesure depuis un an ce dispositif apparaît limitée et que sa mise en oeuvre mérite d'être précisée. Certaines priorités peuvent en revanche surprendre, notamment la majoration exceptionnelle du taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués au au profit des seules associations cultuelles, alors que tant d'autres associations ont besoin d'être soutenues. Enfin, ce projet de loi de finances rectificative est censé organiser une sortie progressive des dispositifs de soutien, prolongés certes par des mesures de relance, mais cette étape devrait marquer la fin du « quoi qu'il en coûte ». Le programme de stabilité présenté en avril dernier par le Gouvernement visait d'ailleurs une réduction de la dépense publique de 60,4 % du PIB en 2021 à 56 % dès 2022, le taux de prélèvements obligatoires restant inchangé. Beaucoup dans la majorité sénatoriale appellent à cette réduction générale de la dépense publique, mais plaident pourtant, par leurs amendements, pour prolonger ou amplifier tel ou tel dispositif budgétaire ou dépense fiscale. Je comprends leurs intentions, tout en notant que, à défaut de réduire la dépense, seules des initiatives sur le volet relatif

à celui-ci toute marge de manoeuvre en recettes, le condamne demain soit à des hausses brutales d'imposition soit à sacrifier des politiques publiques dont on pressent, notamment à la lecture de l'audit réalisé par la Cour des comptes à la demande du Premier ministre, qu'elles concerneraient par priorité le champ social. Pour ma part, je ne m'y résous pas ! La parole

Il n'en contient pas moins un certain nombre de mesures budgétaires et fiscales qui viennent modifier l'équilibre voté en loi de finances initiale. C'est bien le minimum, alors que le contexte sanitaire continue de peser lourdement sur l'ensemble des agents économiques et affecte notre capacité à faire redémarrer une croissance durable. Je remarque d'abord la fragilité persistante des hypothèses macroéconomiques. L'année 2020 a été pour cela tout à fait inédite, avec une chute vertigineuse de l'activité économique, puis un rebond limité en deuxième partie d'année avec la levée, puis malheureusement le retour, à l'automne, des restrictions sanitaires. Les Les quatre lois de finances rectificatives adoptées l'an dernier ont eu pour conséquence des reports importants de crédits sur 2021, ce qui a contribué à repousser la présentation d'un nouveau texte, d'abord annoncé pour le mois de mars. Notre capacité à construire un budget fiable sur le cycle budgétaire est d'autant plus importante que notre économie a aussi besoin de confiance pour pouvoir se projeter. Le décret d'avance de plus de 7 milliards d'euros, un record depuis 1958, vient nuancer ce propos. Le Gouvernement s'était gardé d'en faire usage depuis 2017, et c'était tout à son honneur. On peut dire que cette pratique, parfois controversée, est revenue en force avec la publication, le 19 mai dernier, La réalisation des hypothèses de croissance économique et de solde budgétaire en 2021 dépendra de notre capacité à continuer de maîtriser la pandémie, en particulier une éventuelle quatrième vague dont on voit déjà augmenter le risque de survenue pour l'automne. Le déficit budgétaire de 9,4 % du PIB, légèrement plus élevé qu'en 2020, peut inquiéter. Il s'explique en partie, comme je l'ai dit, par des reports de crédits votés en lois de

Outre la poursuite des dispositifs de soutien existants, les entreprises bénéficieront de davantage de souplesse pour affronter cette période difficile. Les ménages ne sont pas oubliés, avec la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, en particulier pour les salariés de deuxième ligne. Le groupe du RDSE porte, toujours, une attention particulière au secteur agricole et aux territoires ruraux, qui plus est durement touchés par des gelées tardives au printemps. Les dispositions introduites à l'Assemblée nationale sur la dotation pour aléas ou encore le report de la hausse de la taxation du GNR vont dans le bon sens. Nous présenterons des amendements pour aller plus loin dans cette direction. Enfin, les mesures d'aide aux collectivités et surtout aux établissements publics locaux, prévues à l'article 10 du texte, permettront à ces structures et aux collectivités dont elles dépendent de mieux faire face aux pertes de recettes tarifaires, ce qui permettra de combler une lacune du plan de soutien. Je salue également des mesures sectorielles telles que l'aide aux gérants de discothèques, établissements qui ont été contraints de rester fermés depuis le début de la crise sanitaire il y a plus d'un an.

qui jouent un rôle essentiel de maintien du lien social- cette mesure est inspirée de la proposition de loi qu'Éric Gold a déposée en début d'année. Il n'est pas possible de commenter en détail l'ensemble des mesures. Je retiens simplement que ce texte marque la volonté pérenne du Gouvernement de continuer à soutenir l'économie tant que les conséquences des restrictions sanitaires pèseront sur les entreprises- le « quoi qu'il en coûte ». Le coût budgétaire de cet engagement est considérable et il faudra, le moment venu, en tirer les conséquences et faire des propositions. Regrettant peut-être un manque de lissage entre la résolution de la crise et le retour à un rythme normal, ainsi que des mesures proposées par la majorité sénatoriale qui risquent de dégrader encore davantage les comptes, la majorité des membres du groupe du RDSE devrait s'abstenir sur le vote de ce projet de loi de finances rectificative.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis pour la saison 5 du PLFR ! M. Bruno Le Maire a commencé de siffler la fin de la partie. Il pose d'ores et déjà l'acte de décès du « quoi qu'il en coûte ». Le plus inquiétant est que le ministre affiche son obsession sur le sujet de la dette publique comme moyen de remettre en cause encore et toujours notre modèle de protection sociale. Toujours aucune conditionnalité au versement des aides : pourtant, un rapport récent a montré que, sur les vingt-sept groupes du CAC 40 ayant bénéficié de l'activité partielle, seize ont versé des dividendes en 2020 et vingt-deux en 2021. Je cite M. Le Maire : « Ce budget amorce la transition vers un retour à la normale. » C'est un budget de retour à la normale pour une situation qui ne l'est toujours pas : le variant delta fait courir le risque majeur d'un regain de la propagation et du taux d'incidence. En dépit d'une progression de la vaccination, au ralenti aujourd'hui, à peine la moitié des Français ont reçu une injection et moins d'un tiers ont bénéficié de deux doses. Le variant delta semble résister davantage au sérum- c'est l'échappement immunitaire. La sortie de crise est-elle illusoire ? de loi de finances rectificative n'indique que les finances publiques sont mobilisées pour envisager une quatrième vague. Toute la politique du Gouvernement s'inscrit, comme depuis le début, dans une impréparation inquiétante, alors que notre situation nécessite au contraire une planification en amont. Anticiper, prévoir et encore prévoir, c'est le seul moyen pour garantir la protection de la population et l'efficacité des dépenses au premier euro en matière d'urgence et de relance. La crise sanitaire a révélé, même s'il n'est pas l'heure d'en faire le bilan tant qu'elle n'est pas derrière nous, la gestion pour le moins approximative de l'exécutif. On relève notamment près de 10 milliards d'euros de dépenses de santé supplémentaires par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 Des sources gouvernementales indiquaient que le budget de la sécurité sociale présentait « des provisions larges au cas où l'épidémie devrait durer encore longtemps ». Bilan : vous prévoyez 1,5 milliard d'euros pour la campagne de vaccination, soit 3,5 fois moins que son coût actuel chiffré à 5,2 milliards d'euros. La gestion des crédits destinés à renforcer les participations financières de l'État dans la crise sanitaire est notoirement insuffisante. Vous vous en êtes servis comme d'une réserve de crédits que vous avez détournée de son usage initial, en la dépouillant de 16,2 milliards d'euros.

c'est pourtant l'un des outils indispensables à la préservation de l'emploi qui se trouve finalement amputé de 11,4 milliards d'euros. Tels de véritables prestidigitateurs, vous jonglez avec les crédits, quitte à nous en faire perdre la trace, tout comme aux citoyennes et citoyens de ce pays. Les mesures fiscales contenues dans ce texte s'inscrivent dans la philosophie du ministre de l'économie qui assène : « Nous le savons tous, le premier problème de l'économie française est un problème d'offre ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce gouvernement s'emploie avec une extrême vigueur à baisser l'impôt des entreprises. Sa dernière trouvaille : rendre illimitée la possibilité pour les grandes entreprises d'imputer un exercice déficitaire jusqu'à trois années en arrière-

Comme toutes les autres aides publiques versées depuis le début de la crise sanitaire, votre gouvernement qui s'est déjà fait démentir par les grandes multinationales à de nombreuses reprises, notamment sur le non-versement de dividendes, persiste à ne rien exiger en retour des milliards d'euros

Ce collectif budgétaire est en premier lieu l'occasion pour le Gouvernement d'ajuster sa prévision de croissance à un taux de 5 % pour cette année. Cet objectif, jugé réaliste par le Haut Conseil des finances publiques, semble raisonnable, si la main-d'oeuvre est suffisante pour répondre à la demande. Toutefois, c'est un déficit à hauteur de 228 milliards d'euros qui est désormais attendu, alors que la loi de finances initiale votée en décembre l'estimait à 173 milliards. La dette publique se creuse et s'établit dorénavant à 118 % du PIB. La dégradation du solde public est en partie liée au large soutien de l'État à l'économie, soutien auquel notre assemblée a activement contribué l'an passé, tout en maintenant sa vigilance sur la trajectoire budgétaire. Parmi les 20 milliards d'euros de ce texte, 9,8 milliards alloués au plan d'urgence permettent de prolonger le dispositif de chômage partiel, le fonds de solidarité pour les entreprises et la compensation des exonérations de charges. Ce sont également 4,9 milliards d'euros qui sont accordés au titre du plan de relance. Au-delà des importantes « recharges » de crédits, plusieurs mesures doivent retenir notre attention.

Je souhaite saluer l'éligibilité au fonds de solidarité des régies à caractère industriel et commercial, ainsi que la mise en place d'un fonds d'urgence pour les régies à caractère administratif. Cette juste extension du dispositif, à laquelle vous avez ouvert la voie, monsieur le ministre, devant la commission des finances en mai dernier, doit notamment permettre aux régies thermales de supporter le lourd tribut de la crise et de préserver des milliers d'emplois, dont 400, à titre d'exemple, dans mon département, le Jura- je vous en remercie vivement. Par ailleurs, le groupe Union Centriste proposera de maintenir à 2023 le report de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole non routier afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, déjà confrontées à la hausse des prix de certaines matières premières.

afin de ne pas pénaliser les structures intercommunales qui, faisant preuve de volontarisme, ont adopté des pactes financiers et fiscaux avant la suppression envisagée de cette taxe. Notre groupe plaidera également pour un amendement proposant de fiscaliser les aides versées, si le solde du compte de résultat de l'entreprise est supérieur à la moyenne du solde des trois exercices comptables avant la crise, afin de s'assurer de la maîtrise de la dépense publique. Monsieur le ministre, je n'imagine pas que des revenus perçus antérieurement à la crise et soumis à l'impôt puissent être dopés par les aides de l'État et exonérés de fiscalité. Favorable à un soutien réel et justement réparti, le groupe Union Centriste votera, dans sa très grande majorité,

le 23 juin, la Commission européenne a officiellement validé le plan français de relance et de résilience. Les 40 premiers milliards d'euros débloqués par la Commission sur l'enveloppe totale des 100 milliards de notre plan de relance vont doper l'économie et, peu à peu, les milliards longtemps promis vont devenir réalité. Cette annonce marque une étape historique de la construction européenne, mais à plus court terme, elle constitue avant tout une excellente nouvelle pour notre économie. La relance devient effective, parce que son financement le devient aussi. Le projet de loi de finances rectificative dont nous commençons aujourd'hui l'examen acte le rebond de notre économie. En tablant sur une croissance de 5 %, nous avons confiance dans la résilience de nos entreprises et dans le dynamisme de ceux qui peuvent consommer. L'autre bonne nouvelle de ce texte, qui en est le corollaire direct, c'est la fin du « quoi qu'il en coûte » ou du moins le début de la fin du « quoi qu'il en coûte » ... Le Gouvernement a enfin validé ce changement de paradigme. Nous allons progressivement nous défaire du régime des aides généralisées pour lui substituer un régime d'aides ciblées. Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe Les Indépendants a soutenu les mesures de sauvetage et de relance. La puissance publique, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, a été présente aux côtés des entreprises et des particuliers au moment où il le fallait et là où il le fallait. Notre groupe soutient aujourd'hui la sortie progressive du « quoi qu'il en coûte Nous sommes trop attachés à la réduction de l'endettement public pour ne pas nous en féliciter. Le moment choisi semble le bon : d'une part, notre pays s'est enfin engagé sur la voie d'une relance vigoureuse ; d'autre part, la stratégie vaccinale nous laisse espérer une victoire prochaine contre le virus, sous réserve de son parfait déploiement et de mesures de consolidation pour une protection prolongée. Mais cet espoir ne doit pas nous bercer d'illusions, car le dynamisme de la croissance ne saurait cacher la dégradation très inquiétante de nos finances publiques nous contenons à peine le déficit en deçà des 10 % du PIB, les dépenses publiques aspirent plus de 60 % de la richesse créée dans notre pays et la dette a dépassé, au premier trimestre, 118 % du PIB. Il faut encore rappeler ces chiffres, car ils conditionnent notre action. En matière de politique économique, nos décisions doivent permettre à la fois de réinjecter un maximum de liquidités dans l'économie, de stimuler la demande, et de limiter l'impact du soutien sur nos finances publiques. La plupart des mesures de ce texte vont dans le bon sens. Elles s'inscrivent dans la continuité de mesures consensuelles. ainsi de la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou encore de la prolongation des prêts garantis par l'État et du fonds de solidarité. Il en va de même du dispositif de prôné depuis longtemps par le Sénat et enfin retenu par le Gouvernement. Mais le projet de loi n'apporte aucune réponse au grand défi qui se pose à notre économie : comment mieux mobiliser l'épargne des Français pour préparer l'avenir ? Notre groupe a déjà eu l'occasion de présenter une proposition de loi visant à instaurer un dispositif à cette fin, mais le Gouvernement n'a pas jugé cette mesure opportune. Nous ne remettrons pas l'ouvrage sur le métier, car le débat a déjà eu lieu dans cet hémicycle. Pourtant, les conditions qui nous ont conduits à porter une telle mesure n'ont pas évolué : d'une part, la situation de nos finances publiques demeure excessivement dégradée ; d'autre part, l'épargne des Français n'a jamais été aussi importante. Or, puisque nous devons dans un même élan sortir de la crise et investir pour préparer l'avenir, et ce sans dégrader davantage nos finances publiques, mobiliser l'épargne au service de l'économie demeure selon nous une priorité. Nous ferons des propositions dans ce sens, notamment pour renforcer la santé financière de nos petites entreprises et de nos associations. Non, la relance ne passera pas uniquement par un rebond spectaculaire de la consommation. Il ne s'agit pas, bien sûr, de bouder le retour à la vie normale, mais seulement d'être lucides sur les occasions que nous devons saisir pour que la France tienne son rang. Il faudra tout à la fois engager une ambitieuse réduction des dépenses publiques, investir dans les infrastructures, l'innovation technologique et la transition écologique et soutenir le tissu économique et social dans nos territoires. C'est cette équation que nous devons résoudre, si nous voulons que la France soit en mesure de relever les défis de son temps. Ce projet de loi de finances rectificative constitue une bonne première étape en ce sens. La commission des finances a d'ores et déjà fait des propositions très intéressantes pour améliorer les dispositions du texte et surtout mieux territorialiser la relance. Nous les soutiendrons dans leur grande majorité. La parole

la continuité l'approfondissement d'un budget initial que nous avions déjà dénoncé comme étant très largement déséquilibré : tout pour les entreprises, trop peu pour les gens et pas assez pour préparer l'avenir.

soit écologique ou sociale, ni étude d'impact. Pendant ce temps, de grands groupes du CAC 40 qui ont pourtant connu des pertes en 2020 continuent à verser des dividendes

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous voyons chaque jour un peu plus se dessiner la perspective d'une sortie de crise, le projet de loi de finances rectificative est déterminant pour la relance de notre économie. économie. Il est déterminant en raison de ses objectifs, à savoir, d'une part, aider les secteurs les plus sinistrés grâce au rechargement des dispositifs d'urgence et, d'autre part, préparer la sortie de crise en accélérant le plan de relance du Gouvernement. La prévision de croissance du PIB du Gouvernement pour 2021 reste encourageante, puisqu'elle se maintient à hauteur de 5 %. Nous le constatons autour de nous avec soulagement : l'économie repart, et la consommation des Français augmente. Mais ce contexte ne doit pas nous faire perdre de vue les secteurs qui ont été durement touchés et qui continuent de l'être. Si le « quoi qu'il en coûte » a permis de sauver bon nombre d'entreprises et d'emplois, nous devons continuer d'accompagner les secteurs qui font encore face à de nombreuses difficultés. Le Gouvernement s'y engage, puisque ce PLFR recharge considérablement les dispositifs d'urgence dans le contexte de sortie de crise. Il ratifie les modifications introduites par décret d'avance des crédits de 500 millions d'euros supplémentaires pour la prise en charge du chômage partiel, et de 6,7 milliards d'euros au bénéfice du fonds de solidarité, qui sera prolongé jusqu'au 31 août 2021 pour les entreprises. De plus, pour accompagner les entreprises jusqu'au bout de la crise, la date limite d'octroi des prêts garantis par l'État est reportée du 30 juin au 31 décembre 2021. Depuis de nombreux mois, l'État a également apporté la preuve de son soutien sans réserve aux collectivités territoriales les plus touchées par la crise. Songez, mes chers collègues, alors que le déficit de l'État a frôlé les 8 % du PIB en 2020, que les collectivités n'ont connu en moyenne année. Si nous pouvons nous en réjouir, cela ne doit pas pour autant nous conduire à baisser les armes, car ces chiffres recouvrent parfois des disparités dont les conséquences sont bien difficiles à vivre pour les collectivités qui en souffrent. C'est pour cela que l'État et le Gouvernement se mobilisent à nouveau, dans ce budget, pour soutenir les services publics locaux de proximité. L'essentiel du coût de la crise a été supporté par l'État et les organismes de sécurité sociale. Ce PLFR renforce le soutien de l'État grâce au « filet de sécurité » et aux 200 millions d'euros de crédits supplémentaires à destination des collectivités locales. Ces 200 millions d'euros serviront à dédommager les pertes réelles subies par les services publics industriels et commerciaux en régie à la compensation intégrale de la baisse d'épargne brute constatée. Ce dispositif sera complété par un fonds d'urgence destiné à soutenir les collectivités locales lourdement affectées par la crise en raison de l'exploitation des services publics à caractère administratif.

retrouver le chemin de l'équilibre et leur permettre de bénéficier de la hausse du taux de taxe d'habitation qu'elles ont votée en 2018 et 2019 avec le soutien de l'État et des chambres régionales des comptes. Ces communes sont peu nombreuses, mais il est essentiel que nous puissions les accompagner dans leur démarche. Parce que la crise a renforcé les inégalités, le Gouvernement consacre par ailleurs de nouveaux moyens au soutien des secteurs et des publics les plus fragilisés par la crise. Je pense notamment au secteur agricole, qui a subi épisode de gel au mois de mars et une épidémie de grippe aviaire. Ces épreuves difficiles justifient la mise en oeuvre de mesures d'aide à hauteur de 350 millions d'euros. Ce PLFR prévoit par ailleurs l'ouverture de 700 millions d'euros de crédits qui permettront de maintenir 200 000 places d'hébergement d'urgence jusqu'à la fin de l'année. Je pense également au monde du sport- auquel je suis attaché

Industries du futur, 46 millions d'euros de subventions réaffectées au développement de l'avion à hydrogène, 4,2 milliards d'euros supplémentaires pour rembourser les dépenses d'activité partielle covid, 11 milliards d'euros pour renforcer la part verte du plan de relance de mesures budgétaires qui permettront d'accélérer l'exécution du plan de relance au service de la transition énergétique. Accompagner les secteurs sinistrés par des dispositifs d'urgence actualisés tout en soutenant les collectivités, les entreprises

Cela montre qu'on aurait pu faire plus et mieux en 2020- nous y reviendrons d'ailleurs lors de l'examen de la loi de règlement -, mais aussi, que, par un jeu

si la crise sanitaire semble marquer le pas dans notre pays et s'il y a un début de reprise économique, la crise sociale, elle, frappe toujours de plein fouet les plus fragiles de nos concitoyens. À cet égard, monsieur le ministre, force est de constater que le compte n'y est pas. Après quatre ans de recul en matière de justice fiscale, ce projet de loi de finances rectificative ne comporte toujours aucune mesure de rééquilibrage de l'impôt. Avec vous, c'est « quoi qu'il en coûte mais jamais pour les plus aisés de nos concitoyens ! Même le président des États-Unis, qui n'est pas connu pour être un dangereux socialiste, prend des mesures très fortes d'imposition sur les grandes entreprises, tout en reconnaissant que la théorie dite « du ruissellement » n'a jamais fonctionné. En France, après les propositions d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole sur les successions, l'économiste Benoît Coeuré plaidait ce matin dans « pour une augmentation temporaire de la fiscalité qui pourrait porter sur le patrimoine, sur les revenus ou sur les successions ».

fait, la politique de l'offre que vous menez depuis 2017 n'a pas montré une grande efficacité ; elle est restée incomprise des Français, alimentant le sentiment d'injustice sociale. Avec la crise que nous vivons, elle est devenue insensée. Pourquoi vous priver de recettes supplémentaires, alors que le déficit budgétaire se dégradera de près de 50 milliards d'euros, ce qui le portera à 220 milliards d'euros en 2021, et que la dette passera à près de 118 % du PIB ? Alors que la pauvreté explose, que la jeunesse est laissée sur le bord de la route, que les services publics, mis à mal, requièrent plus que jamais le soutien de l'État ? Parce que la solidarité, trop souvent oubliée par l'exécutif, doit retrouver sa place au coeur de nos politiques publiques, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposera de nombreux amendements visant Monsieur le ministre- vous le savez -, ces dix-huit derniers mois, vous nous avez toujours trouvés à vos côtés pour voter en responsabilité les mesures de restriction dues à la crise sanitaire et les dispositifs budgétaires de soutien indispensables. Nous avons toujours proposé des mesures plus justes socialement, chiffrées et financées par une hausse de l'effort de ceux qui le pouvaient. Nous persévérerons dans ce débat, car- nous l'affirmons de nouveau -, les mesures économiques et sociales que vous proposez aujourd'hui ne sont pas suffisantes. De fait, ce budget rectificatif constitue à la fois un minimum indispensable et une nouvelle occasion manquée : pas assez sur le plan d'urgence pour faire face à l'urgence sociale ; pas assez non plus sur le plan de relance, dont chacun constate la mise en oeuvre laborieuse, et qui reste largement absent de ce collectif budgétaire. Vous restez dans un entre-deux et c'est insuffisant, mais également incohérent tant l'évolution de la situation aurait dû vous conduire à bouger davantage les lignes, en recettes comme en dépenses. C'est pourquoi le groupe Socialiste, Écologiste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

-dont vous nous avez saisis seulement quelques jours après que nous nous sommes prononcés sur le décret d'avance portant sur 7,2 milliards d'euros, soit le plafond légal autorisé. Ce PLFR ouvre près de 20 milliards de crédits nouveaux, s'ajoutant aux 28,8 milliards d'euros de crédits de 2020 reportés en 2021 au titre du plan d'urgence, soit autant qu'au cours des douze dernières années.

soit entrée dans les esprits, non seulement de beaucoup de Français, mais aussi des ministres eux-mêmes. Je compatis, monsieur le ministre, à l'idée des arbitrages que vous allez devoir rendre, même si je doute qu'ils entrent dans l'épure des 8 milliards d'euros que nous pouvons peut-être encore nous autoriser. Pour en revenir à ce PLFR, la prévision de croissance retenue par le Gouvernement pour 2021 reste à +5 % ; elle est donc inchangée par rapport à celle figurant dans le programme de stabilité d'avril dernier,

Les données présentées dans ce PLFR témoignent ainsi de la situation très dégradée des finances publiques de la France en 2021. Selon la prévision du projet de loi de finances rectificative, le ratio de dette publique augmenterait de 20 points de PIB entre 2019 et 2021, pour atteindre plus de 117,2 % Alors que le niveau de déficit devrait s'établir en 2021 à un niveau plus élevé qu'en 2020, la résorption du déficit et la soutenabilité des finances publiques constituent les enjeux centraux de la stratégie financière de la France. La trajectoire de rétablissement reste incertaine et, surtout, beaucoup plus lente que dans tous les autres pays européens. Pour la première fois de notre histoire, en 2021, après ce PLFR, le volume des dépenses budgétaires sera plus de deux fois supérieur à celui des recettes nettes, portant le déficit à plus de 220 milliards d'euros. C'est déjà en soi un facteur d'inquiétude majeur, mais après une lecture plus attentive de ce PLFR, la situation semble encore plus préoccupante. Permettez-moi de m'arrêter sur deux points. premier est que ce déficit, bien sûr amplifié par la crise que nous connaissons depuis quinze mois, est en fait structurel. D'une part, la trajectoire de hausse des dépenses publiques depuis le début du quinquennat est très supérieure à nos capacités- une augmentation de 19 milliards d'euros en 2020, et de 41 milliards d'euros en 2021, hors mesures de soutien et de relance.

Notre pays est entré dans cette crise dans une situation moins favorable, plus dégradée que celle de nos voisins européens. Il en sort plus affaibli encore, sans réelle visibilité quant à sa trajectoire. La promesse d'un retour aux 3 % de déficit pour 2027 repose sur le seul pari de la croissance, sans réel engagement en matière de réformes structurelles.

Aussi peut-on s'interroger sur la prolongation des mesures de chômage partiel et sur les 6,3 milliards d'euros que vous proposez d'y accorder au moment même où nous manquons de main-d'oeuvre. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains présentera un amendement tendant à faciliter la participation et l'intéressement dans les petites entreprises une prime de 2 000 euros défiscalisée et désocialisée. Cette mesure vise à maintenir les salariés dans les entreprises, qui connaissent ou ont connu de véritables hémorragies.

Je me réjouis du renforcement du dispositif de report en arrière des déficits, communément appelé. Ce mécanisme comptable et fiscal permet à une entreprise de déduire son déficit actuel de bénéfices antérieurs afin de disposer d'une créance d'impôt sur les sociétés. Permettre le report sur les trois exercices précédents tout en en déplafonnant le montant est une mesure essentielle, que le groupe Les Républicains a défendue l'an passé pour éviter les défaillances d'entreprises en renforçant leur trésorerie. Nous regrettons toutefois de ne pas disposer de réelle visibilité quant au coût de ce dispositif

de ce dispositif pour les entreprises et de ne pas alourdir davantage leurs charges en sortie de crise. Nous vous proposerons par ailleurs une majoration exceptionnelle du taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons à des associations caritatives dans le cadre du dispositif dit Coluche.

Je salue la clarification apportée quant à la possibilité d'effectuer des prêts participatifs, et la prorogation du fonds de solidarité jusqu'au 31 août 2021, une dégressivité de son Je tiens aussi à souligner l'adaptation à la reprise de l'activité des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants que vous proposez. J'en viens enfin aux mesures concernant les collectivités territoriales. Nous saluons la reconduction en 2021 du « filet de sécurité » mis en place en 2020 pour garantir les recettes du bloc communal. La compensation des pertes de recettes pour certaines régies publiques non accompagnées par le dispositif d'activité partielle, que nous vous avions proposée en 2020, est aujourd'hui reprise De même, la mise en place d'une dotation pour certaines collectivités en difficulté répond à une attente. Toutefois, le compte n'y est pas. Dans son rapport annuel, le Comité des finances locales (CFL) évalue l'impact de la crise sanitaire pour les comptes des collectivités locales à 5,5 milliards d'euros être mis en regard des 240 millions d'euros de crédits de sauvegarde financés par l'État l'an passé selon l'estimation du même CFL. je ne peux conclure sur le volet des collectivités sans regretter les lourdeurs constatées sur le terrain dans le cadre de la mise en place du plan de relance : dossiers complexes, exigences parfois contradictoires, délais longs et inadaptés, notamment au titre de la dotation

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, ce premier projet de loi de finances rectificative de 2021 n'est pas moins que le cinquième depuis le début de la crise sanitaire. Tout au long de cette crise, la France- c'est vrai -a su mobiliser un large panel de mesures pour soutenir efficacement les entreprises, leurs salariés

Ces mesures sont certes coûteuses, mais elles sont nécessaires pour maintenir le pays debout et en état de marche au moment où il s'agit de réussir la reprise. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit maintenant réussir l'accompagnement de la sortie de crise, réussir la relance, réussir la transition vers un nouveau modèle de développement se fixant comme objectif la souveraineté de la France et de l'Europe dans les secteurs stratégiques, la préservation de l'environnement, la justice sociale et territoriale. Tels sont les défis d'avenir que notre pays devra absolument relever.

Les dispositifs existants, qui sont réabondés, sont complétés par des mesures bienvenues de soutien ciblées, telles que les aides en faveur des agriculteurs affectés par l'épisode de gel. Le texte prévoit aussi des dispositions que le groupe Union Centriste appelait de ses voeux : l'assouplissement du mécanisme de report en arrière des déficits, la prorogation de la garantie de l'État au titre des PGE,

moduler la prime de pouvoir d'achat en fonction du niveau d'exposition au virus, de façon à reconnaître l'engagement de ceux qui, en première ligne, ont pris des risques pour assurer la continuité des services auprès des Français. S'agissant des pertes de recettes tarifaires, nous vous avions alerté, monsieur le ministre, sur l'inégalité de traitement entre les collectivités gérant leur service en délégation de service public (DSP) et celles qui ont fait le choix de la régie.

communes doivent pouvoir bénéficier de cette compensation. Vous répondez à notre demande au travers de l'article 10 : je tiens à vous en remercier, car c'est une avancée importante. Cependant, les critères d'éligibilité sont trop contraignants lorsqu'il ne s'agit pas de SPIC, et le montant prévu, de 200 millions d'euros, me paraît insuffisant. En conclusion, monsieur le ministre, comme l'a indiqué notre collègue Sylvie Vermeillet, le groupe Union Centriste soutiendra ce texte tout en proposant quelques évolutions, de la même manière que nous avons soutenu la stratégie visant à protéger les Français pendant la crise. Il nous faudra toutefois bâtir sans tarder une stratégie collective de redressement des fonds publics. La parole est à M. Thierry Cozic.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes arrivés au bout de nos dogmes économiques ». Cette phrase, prononcée par le Président de la République au G7 de Biarritz en 2019, laissait poindre un changement de paradigme dans notre approche de l'économie en France.

voie. Si vous n'avez de cesse de traquer les moindres aspérités des plus précaires, les aides pour les plus aisés ne sont conditionnées qu'à la sacro-sainte confiance que vous leur accordez aveuglément Dernièrement, alors que la pandémie de covid-19 n'en finit pas de ne pas finir, et alors que les groupes du CAC 40 continuent de bénéficier d'aides publiques massives, ces derniers ont versé 51 milliards d'euros à leurs actionnaires, soit 22 % de hausse par rapport à l'année passée.

pour les plus précaires, suspicion et flicage sont de mise, pour les plus aisés, confiance et pacte de responsabilité le sont. Chacun appréciera sur qui pèse l'obligation de justification La conditionnalité des aides n'est pas le seul écueil qui semble poindre dans votre politique financière et économique : le plan de relance que vous avez mis en place est déjà obsolète ; il est incomplet et lacunaire.

Pourtant, quand on compare les budgets financiers, il manque un ordre de grandeur : en effet, les Chinois et les Américains font dix fois plus que nous. Il nous faut donc un plan de relance de l'investissement dans une perspective de moyen et de long terme.

Néanmoins, si nous ne voulons pas nous retrouver dès décembre prochain avec un nouveau PLFR, la question de l'accompagnement de sortie de crise est centrale. Je rappelle que l'endettement brut des entreprises non financières a augmenté de 170 milliards d'euros de février à septembre, ce qui constitue une singularité bien française. À cet endettement, il faut de plus ajouter les dettes qui découlent du report du paiement des impôts et des cotisations. Nous devons dès maintenant réfléchir à des critères opérationnels d'annulation sélective de dettes pour éviter les effets d'aubaine. Lorsque cela est possible, une approche au cas par cas est nécessaire pour mettre à contribution non pas seulement l'argent public,

Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de tirer les conséquences politiques des déclarations du Président de la République ? C'est le moment, puisqu'il paraît que nous sommes arrivés « au bout de nos dogmes économiques

Réjouissons-nous que le pays se relève d'une période longue et difficile, que nos entreprises se remettent en ordre de bataille et que l'emploi retrouve du dynamisme. S'il est bon d'être optimiste, il est également de notre responsabilité d'être réalistes. En effet, bien que la croissance semble repartir à la hausse, cette reprise demeure loin de compenser les pertes

finances rectificative pour l'année 2020 ont fait bondir la dette de près de 20 points du PIB, ce qui constituera- je le dis avec certitude -une problématique réelle pour les contribuables, les entreprises et surtout les générations à venir.

en ce qui concerne les intempéries qui ont frappé notre pays en ce début d'année et qui ont occasionné des pertes considérables pour de nombreuses exploitations agricoles. Je veux tout d'abord évoquer l'épisode de gel et ses conséquences pour nos agriculteurs, arboriculteurs et viticulteurs. On se souvient que le Premier ministre s'est rendu dans les territoires touchés en promettant aux exploitants une aide de 1 milliard d'euros pour compenser les pertes, sous forme d'aides directes ou d'exonérations de charges. Ce PLFR aurait dû budgétiser la dépense annoncée. Or tel n'est pas le cas. Seuls 314 milliards d'euros ont été inscrits, dont en réalité 115 milliards sont destinés à l'indemnisation de l'épisode de gel, et 200 milliards sont consacrés aux promesses faites en 2020 concernant la betterave et la grippe aviaire. j'imagine que vous allez nous dire que nous devons attendre le bilan final pour indemniser les exploitants. Cependant, je m'étonne que le Premier ministre puisse annoncer des aides aussi élevées sans avoir mesuré les pertes réelles, et que l'État intervienne de nouveau sur des risques assurables, quitte à créer un doute sur la nécessité de s'assurer ou pas,

Pour rappel, le prix a été fixé contractuellement pendant vingt ans à 60 centimes, et sur une décision de votre gouvernement dans le dernier projet de loi de finances, il est passé à 2 centimes. Cette baisse conduira de nombreuses exploitations agricoles, qui ont investi dans cette énergie renouvelable, à la faillite. Comment l'État peut-il s'autoriser ainsi à ne pas respecter ses engagements contractuels ? Décidément, les annonces ne sont pas budgétisées et les contrats ne sont pas honorés ! On ne s'étonnera donc plus du manque de confiance des Français dans la parole des politiques. soulève donc plusieurs questionnements relatifs à l'agriculture, et nous serions bien évidemment rassurés de vous entendre sur ces deux points, qui apparaissent incontournables dans l'examen de ce texte au Sénat. Nous attendons du Gouvernement une rigueur dans la tenue de ses engagements, et des éclaircissements sur des points qui demeurent incertains. La

sont épuisés, ou plutôt auraient été épuisés, depuis le début de cette semaine. Le décret d'avance nous permet donc de faire face aux engagements pris et d'apporter aux entreprises et aux bénéficiaires de ces aides les fonds nécessaires, sans qu'il y ait de rupture.

par le cycle normal du travail des assemblées, et par un certain nombre d'échéances et de textes en discussion. Nous espérons une adoption définitive du texte d'ici au 21 juillet prochain. Ce décalage

nous avions retenu l'hypothèse, non pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un strict point de vue budgétaire, d'un confinement de deux mois plutôt que d'un seul mois. Même si nous souhaitions l'inverse, nous savions que nous n'aurions pas d'autre possibilité d'abonder les crédits. Il valait donc mieux être prudent et prévoir le pire pour pouvoir y faire face.

aux engagements relatifs à certains phénomènes comme la grippe aviaire ou la jaunisse de la betterave, mais aussi à une première tranche d'indemnisation pour les agriculteurs victimes du gel. Nous savons, en effet, que les conséquences de cet épisode de gel sur la trésorerie et le revenu des agriculteurs vont intervenir au rythme des récoltes, et selon une saisonnalité particulière, que nous suivons. Je puis vous assurer que, comme ministre en charge des comptes publics, je suis particulièrement « comptable », si vous me permettez l'expression, des engagements pris par le Premier ministre, et que ceux-ci seront tenus. Ils le seront à hauteur de 1 milliard d'euros, grâce à la mobilisation du dispositif d'exonérations,

50 milliards d'euros de décaissements, puisque, bien évidemment, en matière de subventions aux collectivités, comme dans d'autres domaines, il y a un délai entre la mobilisation des crédits sous forme d'engagements et leur décaissement à réalisation, après parfois quelques procédures.

est importante. La Commission européenne et l'OCDE considèrent que le taux de croissance de la France sera le plus élevé de la zone euro, à hauteur respectivement de 5,7 % et 5,8 %. Nous avons fait le choix « prudent

rester fidèles à notre ligne d'extinction progressive des mesures d'urgence. Le Premier ministre a précisé, le 10 mai dernier, les conditions dans lesquelles le fonds de solidarité allait être progressivement éteint : la prise en charge différentielle du chiffre d'affaires avec un caractère dégressif, ou la remontée à un niveau un peu plus important du reste à charge pour les employeurs, en matière d'activité partielle, et l'orientation des secteurs qui en ont le plus besoin vers l'activité partielle de longue durée. Cet objectif est

Je ne vois pas comment les Français peuvent comprendre quelque chose aux finances publiques, si on leur parle toujours d'équilibre, alors que les finances sont totalement déséquilibrées. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat ! Je pense donc qu'il faut plutôt parler des « conditions générales du déséquilibre financier

dont on essaye de définir les conditions générales dans cette première partie du texte, il faudrait diviser les dépenses publiques par deux. Ce n'est pas ce que je demande, mais c'est ce qu'il faudrait faire pour arriver à l'équilibre. Il faudrait supprimer toutes les missions, « Enseignement scolaire », « Recherche et enseignement supérieur

Il s'agit d'une mesure simple à mettre en place, qui pourrait bénéficier immédiatement aux 4,5 millions de Français qui l'utilisent. C'est pourquoi, cet amendement vise à faire passer le plafond d'exonération de 5,55 euros à 7,50 euros. C'est un soutien bienvenu, alors que le secteur de la restauration a subi deux longues périodes de fermeture administrative, et voit son activité encore fortement réduite par les jauges imposées par la situation sanitaire jusqu'à aujourd'hui. Le titre-restaurant est un outil souple et performant pour agir sur le revenu net disponible,

M. Claude Nougein. Le présent amendement vise à revaloriser la valeur faciale des titres-restaurants, dans le double objectif d'accroître le pouvoir d'achat des 4,3 millions de salariés qui en bénéficient, et de soutenir le secteur de la restauration, durement éprouvé dans le contexte de la crise sanitaire. En pratique, cet amendement tend à relever le plafond d'exonération de l'impôt sur le revenu de la contribution patronale de 5,55 euros à 7,50 euros, ce qui permettrait aux entreprises qui le souhaitent de porter la valeur maximale du titre-restaurant à 15 euros, contre 11,10 euros actuellement. La revalorisation du titre-restaurant constituerait ainsi un outil efficace de relance de l'économie. En outre, d'un point de vue budgétaire, cette mesure présente un caractère vertueux, puisqu'elle s'accompagnerait d'une augmentation des recettes fiscales assises sur la consommation de biens alimentaires, au premier rang duquel figure la TVA. En parallèle, il convient de veiller à ce que les salariés soient en mesure d'écouler les titres-restaurants qui n'ont pas pu être utilisés jusqu'à présent, en raison des mesures sanitaires. À cet effet, le relèvement du plafond de paiement en tickets-restaurants, actuellement limité à 38 euros par jour dans les restaurants, constituerait une mesure constituerait une mesure particulièrement opportune. De la même manière, il serait souhaitable que le Gouvernement autorise les salariés à utiliser leurs titres-restaurants de 2020 jusqu'à la fin de l'année 2021, ou à échanger les titres-restaurants non utilisés en 2020 et 2021 contre des titres-restaurants émis pour l'année civile 2022.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements, dans la mesure où la hausse du montant exonéré d'impôt sur le revenu pour le salarié ne garantit pas une augmentation, dans les mêmes proportions, de la contribution patronale de l'employeur, ni même un effet positif significatif sur le pouvoir d'achat des ménages. L'employeur détermine, en effet, librement le montant la valeur libératoire des titres-restaurants qu'il octroie au personnel. Pour ces raisons, nous sommes défavorables aux deux amendements.

Le Gouvernement reprend à son compte le dogme qui organise la baisse des recettes de l'État et le démantèlement des services publics, par voie de conséquence. Le niveau de l'impôt sur les sociétés connaît une inexorable décrue. Jusqu'au milieu des années 1980, les bénéfices d'entreprise étaient en effet taxés à 50 %, soit deux fois plus que le taux qui s'appliquera l'année prochaine. Nous étions loin d'une France en première ligne d'un supposé matraquage fiscal,

La presse rapporte à juste titre que les géants des groupes numériques ne s'y sont pas trompés : curieusement, tous ont accueilli avec satisfaction les annonces du G7 Finances. Par exemple, M. Nick Clegg, dont chacun se souvient qu'il est aujourd'hui vice-président des affaires publiques du groupe Facebook,

au-delà de ce que prévoit déjà le dispositif proposé. En effet, les créances de peuvent d'ores et déjà être mobilisées auprès d'établissements de crédit par voie de cession Dailly.

qui, par leur dimension, sont exclues du bénéfice de certaines aides ou assujetties à des plafonds beaucoup trop bas pour que les aides soient véritablement pertinentes. Il s'agit donc, par ce déplafonnement, d'aider certaines ETI ayant pu afficher des pertes de quelques dizaines de millions d'euros au cours de l'année dernière,

Cet amendement a trait au régime fiscal de certaines aides versées aux entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire. Nous connaissons les règles applicables au fonds de solidarité.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé ». Dès sa création en 2005, celle-ci a suscité de fortes contestations. L'objectif était de retenir et d'attirer des holdings en France, en France, une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale pourtant décriée unanimement. De grandes entreprises ont bénéficié de cette niche. Ainsi, en 2007, Danone a économisé 500 millions d'euros d'impôt sur les sociétés sur la cession de Danone Biscuits. En 2009, la niche a bénéficié à 6 200 entreprises et seulement 10 entreprises, à elles seules, ont capté 44 % des coûts du dispositif.

estimation à 5 milliards d'euros par an a été avancée par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui plus qu'hier, compte tenu de la crise économique et sociale, nous ne pouvons plus nous passer de telles recettes pour conduire une action publique proportionnée et efficace.

d'opérations qui font partie de la vie économique d'un groupe d'entreprises. Je vous renvoie, mes chers collègues, à ce qu'en disait le Conseil des prélèvements obligatoires en 2017

nous faisons croître de 38 120 euros à 50 000 euros la fraction de bénéfices des PME imposable au taux réduit de 15 %.

un dispositif de déduction fiscale pour le capital à risque, afin d'aider les entreprises et les inciter à renforcer rapidement leurs fonds propres dans la période de sortie de crise.

Fort de ces observations, je m'en remets à la sagesse du Sénat. de simple évolution du niveau d'une activité qui ne serait l'objet ni d'un abandon ni d'une adjonction n'a pas d'incidence sur les déficits reportables. Les changements d'activité qui emportent des conséquences sur les déficits sont très peu nombreux, comme en témoignent les demandes d'agrément déposées en 2020, soit moins d'une dizaine.

de « simplification »- vous la présentez comme telle -, nous nous priverions de capacités de contrôle et de garde-fous. Le maintien d'emplois en contrepartie du maintien des déficits serait contraire à la politique de sauvegarde des emplois dans les entreprises rencontrant des difficultés.

aujourd'hui, les entreprises sont invitées à relocaliser leur activité et à s'adapter à l'économie, qui a été modifiée par la crise que nous venons de vivre.

de 1991 à 2011, à savoir la possibilité temporaire d'amortissement accéléré des matériels destinés à économiser

cet amendement vise à prévoir une modalité dérogatoire d'imputation de l'avantage fiscal issu de ce mécanisme d'amortissement, afin de permettre aux entreprises constatant un déficit en raison de la situation économique actuelle de le monétiser immédiatement.

l'initiative américaine en matière d'imposition minimale et de réouverture des discussions sur la taxe numérique, autant je suis interpellé par votre volonté de présenter la politique fiscale américaine comme un modèle de solidarité.

porterait le taux américain à un niveau bien inférieur au taux de 25 % que nous proposons. En matière de fiscalité des particuliers, si nous voulions nous aligner sur un modèle assez proche de celui qui est pratiqué

en conformité avec le droit de l'Union européenne et la jurisprudence administrative le prélèvement prévu à l'article 244 B du code général des impôts, applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu'à certaines distributions réalisés soit par une personne physique non domiciliée en France, soit par une personne morale dont le siège social est situé hors de France.

il est prévu que le nouveau dispositif s'applique aux cessions ou au rachat de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021- à la date d'aujourd'hui

: La parole est à M. Michel Savin. Les établissements sportifs couverts et marchands, notamment les salles de sport, comptent parmi les structures les plus durement touchées par la crise sanitaire.

L'objectif du Gouvernement était d'assurer la neutralité fiscale et sociale des aides versées par le fonds de solidarité. Cette mesure, utile et attendue, compte tenu de l'urgence de la situation, dans certains cas à ce que les entreprises bénéficiaires enregistrent des résultats supérieurs à ceux qu'elles avaient pu enregistrer avant l'apparition de l'épidémie de covid-19. Si elles sont justifiées et légitimes dès lors qu'elles permettent de maintenir à flot les entreprises et d'assurer leur pérennité, les subventions versées au titre du fonds de solidarité ne doivent pas conduire à une sur-indemnisation aux frais des contribuables et des générations futures. Pour garantir pleinement l'équilibre et la justice du Fonds de solidarité pour les entreprises, le présent amendement vise à rectifier le tir, en soumettant à prélèvements obligatoires les aides

n'a pas été bien calibré. Surtout, sur le plan fiscal, il a entraîné des effets d'aubaine extraordinaires. J'en ai constaté chez des chauffeurs de taxi

qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. » Il est minuit. En conséquence, je constate que la session ordinaire de 2020-2021 est close.